n° II-627 rectifié . La loi permet aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de bénéficier d'une recette pour la mise en oeuvre des schémas d'aménagement de gestion des eaux. Elle est constituée par la majoration d'une redevance prélevée par les agences de l'eau. Malgré plusieurs demandes émanant de divers territoires, malgré plusieurs dossiers en cours, cette majoration de redevance n'a jamais pu être mobilisée, et ce alors que le besoin d'autofinancement pour poursuivre les missions des EPTB s'accroît. Est en cause la baisse des contributions des différents financeurs, et notamment des départements. En effet, après arbitrage du Gouvernement, cette recette a été incluse dans les recettes des agences de l'eau, qui sont plafonnées. Par conséquent, la mise en place de la majoration de redevance grèverait les autres bénéficiaires, ce qui entraînerait un conflit d'intérêts sur les territoires. Or des études juridiques montrent que la recette n'entre pas dans les recettes plafonnées des agences, puisque le plafonnement s'applique aux recettes qui bénéficient aux agences. cet amendement, il s'agit d'indiquer clairement que la recette produite par la majoration de redevance est exclue du plafond des recettes des agences de l'eau, définies dans l'article 46 de la loi de finances 2012, et ce au même titre que d'autres dépenses, notamment les reversions à l'Agence française pour la biodiversité

Les établissements publics territoriaux de bassin sont des acteurs essentiels de la gestion de l'eau, le Gouvernement en est parfaitement d'accord. Toutefois, je le rappelle, ils disposent d'ores et déjà de divers financements possibles pour leur action,

L'instauration d'un plafond de recettes pour les agences de l'eau permettant de garantir le respect des objectifs de maîtrise des dépenses publiques et de limitation de la pression fiscale sur les entreprises et les ménages constitue un enjeu important. La mise hors plafond de la sur-redevance EPTB reviendrait au contraire à remettre en cause l'effectivité de ce plafond. La nature des missions financées en partie par cette sur-redevance EPTB locale, et par ailleurs finançables par d'autres biais, ne justifie pas, contrairement au plan Écophyto national, qu'elle soit mise hors plafond des agences de l'eau. Enfin, il convient de rappeler que d'autres acteurs de l'eau, les syndicats mixtes que sont les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (Épage) exercent des missions comparables, voire identiques, sur d'autres territoires, sans bénéficier de l'avantage que serait la mise hors plafond de cette sur-redevance. Pour toutes ces raisons, je demande

Quel est l'avis du Gouvernement ? Ce n'est pas tout à fait la simple suppression d'un Il s'agit de rendre obligatoires la télédéclaration et le télépaiement dès le 1avril 2020 pour les redevables de taxes aéronautiques. Sur le fond, c'est le sens de l'histoire d'aller vers ce dispositif.

des redevables ne sont pas établis dans l'Union européenne. Ces compagnies devront désigner contractuellement un représentant fiscal chargé d'assurer, pour leur compte, le paiement par voie électronique. Pour cette raison très pragmatique,

Concernant les aviseurs fiscaux, nous souhaitons introduire un critère de manquement à caractère international, pour l'extension du régime des aviseurs fiscaux à des problématiques de TVA. Quel est l'avis du Gouvernement ?

En effet, par cet article, il s'agit d'intégrer le régime des SIIC dans la réglementation des aviseurs fiscaux, en raison de l'existence supposée de fraude fiscale, notamment une suspicion de détention d'actions de SIIC par des structures étrangères. Or il existe déjà une retenue à la source de 15 % à 30 %, et les sociétés cotées sont déjà contrôlées par de nombreuses autorités. Par

Des garanties suffisantes doivent donc être prévues. Le dispositif actuel offre les garanties requises, dès lors que les demandes d'accès sont validées par un notaire, officier ministériel appartenant à une profession réglementée. Tel n'est pas le cas des généalogistes. L'extension proposée porterait une atteinte disproportionnée au secret de la vie privée.

maintenu ? La loi Eckert de 2014 a élargi les cas de règlement de succession. Dans ce cadre, il est nécessaire que les généalogistes professionnels puissent diligenter toutes les recherches pour identifier des ayants droit, et pas uniquement sur mandat de notaire, ce qui est extrêmement restrictif.

C'est de la rédaction approfondie ! Cet amendement vise à donner une définition du jaune budgétaire, mais la notion d'effort financier de l'État dans les domaines d'intervention auxquels il se réfère est trop restrictive pour couvrir le périmètre de l'ensemble des jaunes, qui peuvent définir des informations relatives aux actions menées, par exemple, par des opérateurs de l'État. Ainsi, le jaune des agences de l'eau

La reprise de la trajectoire carbone, à laquelle le Gouvernement a dû renoncer l'année passée sous l'effet de la contestation sociale, n'est pas exclue, puisqu'elle fait l'objet d'un débat au sein de la Convention citoyenne pour le climat. telle éventualité suscite de fortes inquiétudes chez les ménages, notamment les plus modestes et ceux vivant en zone rurale, dont le budget « énergie » est de 3 850 euros par an, selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires Selon ce rapport, il existe clairement un déficit d'information dans ce domaine. Il précise ainsi que « le lecteur de la loi fiscale est incapable d'identifier la fiscalité carbone ». Le présent amendement prévoit donc que toute évolution envisagée par le Gouvernement en matière de fiscalité carbone fasse l'objet d'une analyse détaillée quant à son impact sur les ménages et les entreprises, dans le cadre du rapport annuel sur l'impact environnemental du budget institué par le présent article. Une telle évaluation permettra de renforcer l'information du Parlement et des citoyens sur la fiscalité carbone. Elle incitera le Gouvernement à évaluer et à justifier sa politique, afin d'éviter une réforme mal évaluée et mal calibrée, comme celle de l'an dernier. Quel

un certain nombre d'éléments sont communiqués au Parlement en appui des trajectoires plus largement fiscales qui sont décidées. L'article 59 du projet de loi de finances pour 2020 remplace le rapport dédié au financement de la transition écologique par un rapport annuel sur l'impact environnemental du budget. La fiscalité écologique a fait l'objet d'un rapport spécifique, intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat », qui est annexé au projet de loi de finances pour 2020 et a été publié, pour la première fois, le 11 octobre 2019. Enfin, les taxes concernées, leur finalité, l'utilisation des recettes correspondantes, continueront à être présentées chaque année, en toute transparence, de façon aussi détaillée que possible.

à l'atteinte des objectifs de notre politique énergétique nationale, désormais fixés par le législateur dans le cadre d'une « loi quinquennale ». Or, tel qu'il est rédigé, l'article 59 conduira à l'abrogation de cette disposition, qui vient à peine d'entrer en vigueur depuis la promulgation de la loi précitée par le président de la République. C'est regrettable, tant sur le plan de l'information des parlementaires que sur celui de la stabilité des normes. Il n'est pas pensable

Nous avons, commune aux deux assemblées, une délégation au renseignement, pour les sujets très confidentiels liés à la défense et aux services de renseignement.

Le Parlement européen vient de déclarer l'état d'urgence climatique, le 28 novembre dernier, et le programme environnemental de l'ONU vient de lancer un énième cri d'alarme, quelques jours avant la réunion de tous les pays du monde, à Madrid, pour la COP25 sur l'avenir du climat. Les Français sont chaque jour plus sensibilisés à l'impact climatique et sanitaire de l'économie carbonée. Ils se disent prêts à privilégier l'investissement durable, respectueux des ressources planétaires et de l'environnement. Ils n'ont besoin ni de déclaration ni de cri d'alarme ; ils ont besoin d'un signal fort pour retrouver confiance dans une gestion de la crise écologique par les États. Mais où trouver la ressource budgétaire dans un contexte d'endettement structurel ? Une mobilisation de l'effort national est possible. C'est tout l'objet du dispositif In Globo, au coeur de cet amendement proposé par Michel Canevet : favoriser le transfert de l'épargne vers des contrats d'assurance vie individuels ayant un fort contenu écologique. Ainsi, et ainsi seulement, peuvent être palliées les conséquences écologiques- donc, à terme, économiques et humaines désastreuses -d'une gestion trop passive de l'épargne face aux défis des temps présents. L'attractivité des contrats In Globo- ne nous mentons pas -sera nominalement moindre que certaines gestions financières toxiques et court-termistes. Mais elle sera réellement plus efficiente, car il est indispensable que l'épargne responsable s'inscrive dans la longue durée et intègre le développement durable. L'État y contribue en apportant la garantie publique à cette épargne exemplaire, une garantie hors bilan. Le FMI, l'OCDE et l'ONU voient aujourd'hui dans la garantie publique l'outil incontournable pour remédier à un signal-prix du carbone défaillant- défaillant car socialement délicat à mettre en oeuvre, comme nous l'expérimentons depuis plus d'un an. Pour favoriser l'innovation bas-carbone, l'ONU invite les gouvernements à mener des politiques de long terme, permettant de mobiliser les financements privés. Tel est l'objectif central du projet In Globo, qui pourra servir de modèle dans d'autres pays, et d'abord en Allemagne, où l'assurance vie est aussi confrontée à des taux négatifs.

La loi Pacte prévoit déjà des mesures pour développer la finance verte par le biais de l'assurance vie, en introduisant une obligation de présentation d'unités de compte socialement responsables, solidaires et vertes, et en demandant la transparence sur ces unités de compte, clause nécessaire tant il est facile de rendre « vert » un contrat d'assurance vie

des placements financiers et de l'épargne. À ce titre, je trouverais intéressant que le Sénat exprime sa volonté d'un verdissement de l'épargne. J'appelle nos collègues à voter l'amendement de Michel Canevet.

est l'avis du Gouvernement ? L'article 60 du projet de loi prévoit, à compter du 1 janvier 2022, que le paiement en déduction simultanée de la TVA à l'importation auprès de la DGFiP ne sera plus un régime optionnel, mais de droit commun. En conséquence, les entreprises n'auront plus de formalité à effectuer ni d'option à exercer pour bénéficier de ce dispositif. Il n'y a donc pas lieu de préciser, comme le proposent les auteurs de l'amendement, que ce régime, qui sera le régime de droit commun, s'appliquera pour l'ensemble des opérations après notification à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Une telle proposition est, sur le fond, satisfaite, car l'ensemble des opérations bénéficieront du nouveau régime sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire.

en matière de droits d'accise. Cette modification permettra en particulier de s'assurer du maintien des taux de TVA applicables, dans le contexte de la décision du 4 mai 2018 du Conseil d'État. À cette fin, nous proposons également de répéter, au niveau de la loi, l'exclusion du taux réduit pour les boissons alcooliques fournies par les cantines d'entreprises. Ainsi, les boissons autres que les bières de malt, panachés et autres mélanges de bières de malt resteront éligibles

aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires, dispositions qui, pour l'essentiel, n'ont pas été modifiées depuis 1968 et se réfèrent à des notions qui ne correspondent plus à celles qui sont utilisées au niveau national et au niveau européen pour encadrer la production et la commercialisation de ces produits.

conseil. C'est la douane qui mesure au quotidien les activités d'importation et d'exportation, et leurs effets sur la balance commerciale.

ne justifient pas un tel bouleversement, qui ira de toute façon à l'encontre des intérêts des entreprises françaises.

concertée entre deux administrations ayant prouvé leur efficacité : les douanes, d'un côté, la direction générale des finances publiques, de l'autre. Je suis donc défavorable à ces quatre amendements

abondé par le relèvement de cette taxe. Le taux maximum de cette taxe passera ainsi de 0,3 %- 0,2 % pour un produit de biocontrôle -à 3,5 %. Il n'apparaît pas pertinent de conserver la compétence de recouvrement de cette taxe à l'Anses. En effet, il n'est pas opportun que cette agence, chargée d'évaluer et d'autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit, dans le même temps, chargée de recouvrer une recette pour le fonds d'indemnisation nouvellement créé. En outre, l'agent comptable de l'Anses ne dispose pas de leviers de contrôle suffisant. C'est pourquoi il est proposé de confier le recouvrement de cette taxe à la DGFiP, qui assure déjà le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires. Une telle évolution serait parfaitement cohérente avec l'unification des modalités de recouvrement projet de loi de finances. L'affectation de la taxe resterait naturellement inchangée. Afin de permettre la mise en oeuvre de ce transfert dans les meilleures conditions, il est proposé une entrée en vigueur au 1 janvier 2021.

La mission interministérielle France Recouvrement s'est rapprochée de l'Anses pour étudier les modalités de ce transfert, tout en intégrant dans un calendrier une réflexion globale sur les transferts à la DGFiP, voire intégralement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), du recouvrement des prélèvements obligatoires, droits et autres redevances aujourd'hui perçus par les opérateurs. Pour tenir compte des travaux d'ores et déjà engagés et sécuriser le transfert du recouvrement de cette taxe à la DGFiP, il est proposé de n'envisager formellement un tel transfert qu'une fois les analyses complémentaires conduites avec l'Anses, en lien avec la DGFiP.

compensé par une fiscalité locale, l'octroi de mer, qui frappe les importations, sauf exonérations décidées par la collectivité pour des raisons historiquement importantes.

Actuellement, pour être exonérés de droits d'accises sur l'alcool, ces professionnels doivent faire une demande auprès de la douane et déposer une déclaration préalable de profession. Nous proposons de supprimer cette déclaration d'utilisateur pour les professionnels souhaitant bénéficier d'une exonération d'accises sur les alcools dits « dénaturés ».

Sur ce sujet très technique des droits concernant l'alcool et les produits alcooliques tels que le vinaigre ou certains médicaments, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement ?

: La parole est à Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement a pour objet, dans le contexte de la croissance du commerce en ligne, dont on parle régulièrement, de simplifier les formalités administratives liées à la vente à distance de produits soumis à accises. La complexité de la réglementation actuelle en matière de vente à distance de produits soumis à accises dissuade un grand nombre d'opérateurs de développer cette activité ; d'autres s'affranchissent de la réglementation et vendent leurs produits sans acquitter les droits d'accises en France, ce qui entraîne une perte de recettes fiscales pour l'État. Afin de remédier à ces difficultés, les aménagements suivants pour les ventes à distance depuis la France vers l'étranger, la demande de remboursement de l'impôt français pourrait désormais être présentée postérieurement à l'expédition des produits ; pour les ventes à distance depuis l'étranger vers la France, les déclarations et le paiement pourront être globalisés mensuellement, plutôt que réalisées opération par opération, et le système de cautionnement par opération sera remplacé par un agrément pérenne s'appuyant sur une caution solidaire. Dans tous les cas, ces biens pourront être transportés sous couvert de documents commerciaux, sous réserve de comporter les mentions définies par l'administration. Il s'agit en réalité d'une mesure de simplification pour pouvoir

peuvent, sous certaines conditions, être affranchies des formalités administratives à la circulation. Jusqu'à maintenant, les vins sont exclus de ce régime, sauf en cas de déménagement. Cela signifie concrètement que lorsqu'un particulier achète des vins chez un vigneron ou sur un salon, il faut réaliser ces formalités de circulation. Cela joue donc comme un frein administratif dans la commercialisation des produits. Cet amendement vise donc à faciliter ce régime de la vente au particulier en permettant aux vins de bénéficier de cette simplification des formalités de circulation, en supprimant le second alinéa du 9 de l'article 458

les démarches pour la circulation d'essences de parfumerie. Nous parlons ici de produits qui ne contiennent pas d'alcool, mais qui en France sont soumis aux mêmes obligations déclaratives que des produits contenant de l'alcool et encadrés par le code de la santé publique. Ces obligations pour des produits non alcoolisés ne se justifient plus dans le cadre du marché commun. C'est une mesure de bon sens.

comme c'était le cas depuis 2015. Il est à noter que, hormis Aéroports de Paris, aucun exploitant d'aéroport n'a financé ou ne prévoit de financer la mise en service de sas Parafe au moyen

je vous invite à soutenir mon amendement.

En effet, la clause de francophonie, qui constitue un formidable effet de levier en faveur de la production phonographique de talents francophones dans leur diversité, permet de rendre éligible au CIPP l'ensemble des albums de nouveaux talents produits par l'entreprise si au moins la moitié d'entre eux sont des albums d'expression française. Or cette clause est difficile à respecter pour les micro-entreprises qui produisent un nombre très limité de projets par an et qui, en conséquence, privilégient majoritairement les albums en langue anglaise.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement est, bien entendu, attaché à soutenir les petits producteurs de l'industrie phonographique, qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le point de difficulté est le lien de causalité entre la taille de l'entreprise et sa capacité à remplir la condition de francophonie, qui pourrait être contesté au regard d'une rupture du principe d'égalité.

qui est actuellement de 65 % par passager en transit, afin d'alléger la fiscalité des plateformes aéroportuaires françaises défavorisées par rapport à leurs concurrentes européennes nettement moins taxées. Il faut souligner que, depuis 2016, les passagers en correspondance sont déjà exonérés de la taxe d'aviation civile. Il s'agit, par cet amendement, de renforcer la compétitivité, mais aussi l'attractivité des plateformes aéroportuaires françaises, notamment Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly, mais aussi Lyon-Saint-Exupéry, par rapport aux autres plateformes européennes, qui disposent de taxes aéroportuaires très faibles et notoirement inférieures à celles pratiquées en France. Cette exonération permettrait ainsi de mettre à niveau les taxes aéroportuaires françaises avec celles des aéroports européens concurrents. Dans la mesure où la taxe d'aéroport sert à financer les opérations de sécurité et de sûreté, son exonération totale pour les passagers en correspondance se justifie par le fait que la majorité de ces passagers est issue de l'espace Schengen ou d'États comme les États-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne, et bénéficie donc de l'inspection filtrage unique Cet amendement, proposition portée par la quasi-totalité des acteurs du transport aérien dans le cadre des Assises nationales du transport aérien, est une mesure de compétitivité qui permettrait aux compagnies aériennes françaises de développer leur trafic de passagers en correspondance et, ainsi, de gagner en compétitivité par rapport à leurs concurrentes étrangères.

De plus, les coûts liés à la sécurité, comme les moyens d'intervention et de lutte contre les incendies au décollage et à l'atterrissage, continuent d'être acquittés par ces passagers en correspondance, puisqu'ils sont également concernés. L'avis est donc défavorable. Monsieur

Selon une étude récente du Commissariat général au développement durable, 45 % à 60 % du coût total du transport collectif urbain est pris en charge par les entreprises : en plus du versement transport dont elles doivent s'acquitter, soit près de 8 milliards d'euros en 2017, elles participent à hauteur de 50 % au titre de transport mensuel des salariés, pour un montant de 900 millions d'euros. Par ailleurs, la baisse continue durant plusieurs années de la part prise en charge par les usagers fragilise le modèle économique des transports en commun. Les petits réseaux ne sont financés par les usagers qu'à hauteur de 12 % du coût total. Cela a pour conséquence d'alourdir les charges financières des entreprises en matière de financement des transports en commun. Aussi, de telles disproportions ont finalement conduit certaines autorités organisatrices à mener des expériences de gratuité, observées dans une trentaine de réseaux de transport en France. Toutefois, la gratuité totale des transports ne saurait constituer une solution pérenne, car le coût d'une telle mesure serait supporté, pour l'essentiel, par l'entreprise contribuable. En outre, elle fragilise le modèle économique des transports en commun, qui nécessitent davantage d'investissements pour désengorger les zones urbanisées et améliorer ainsi la qualité du service public. Afin d'inciter les autorités organisatrices de la mobilité à ne pas mettre en place une telle mesure, cet amendement proposé par notre collègue René Danesi vise à diminuer le taux du versement transport (VT), lorsque l'autorité organisatrice décide de mettre en oeuvre la gratuité totale des transports. Quel est l'avis de la commission ?

monsieur le sénateur, M. Francis Rol-Tanguy a été missionné par Mme Élisabeth Borne pour produire un rapport proposant une stratégie d'aménagement et de développement durable.

une notion très précise des emplois qui allaient être créés et des taxes qui pouvaient revenir aux diverses collectivités. Tout cela est sur la table ! Je comprends que le Gouvernement puisse être embarrassé d'avoir à rendre ces éléments publics et de faire les additions correspondant à ce que perdra notre département dans cette affaire.

contrasté sur l'impact économique de ce projet pour le Val-d'Oise et la petite couronne. Nous proposons d'avancer en regardant devant nous,

Monsieur le rapporteur général,

en mettant fin à l'écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les grandes plateformes de vidéo à la demande par abonnement, tout en garantissant des ressources stables et pérennes pour le CNC. cet article omet de distinguer le cas des services de vidéo à la demande (SVOD) à l'acte, qui relèvent d'un modèle économique totalement différent de celui de la vidéo à la demande par abonnement. En effet, la hausse du taux de TSV, faite pour accroître la charge fiscale des opérateurs de SVOD, a pour effet collatéral de pénaliser une autre catégorie d'assujettis qui relèvent pourtant d'un marché qui ne connaît ni la même dynamique ni la même structuration. La vidéo à l'acte, et non par abonnement, louée ou achetée, est également redevable de la TSV, mais constitue l'équivalent numérique de la location et de l'achat de DVD. Elle est d'ailleurs alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias. Afin d'éviter que le passage de 2 à 5,15 % du taux de TSV n'aggrave encore les difficultés économiques du marché de la VOD à l'acte, qui connaît une décroissance continue, le présent amendement rétablit la cohérence du dispositif, en étendant l'abattement prévu par le projet de loi pour la vidéo physique aux services de vidéo à la demande à l'acte, dans un principe de neutralité technologique du traitement fiscal. Le régime des plateformes de vidéo à la demande par abonnement reste par ailleurs inchangé.

Cette contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés avait vocation à être répercutée sur les industriels du tabac, mais la pratique a montré qu'elle reposait exclusivement sur le distributeur, et non sur les fabricants. Cet amendement vise à remplacer cette contribution par une augmentation des droits de consommation sur les produits du tabac. Il ne s'agit pas de baisser l'imposition, mais de remplacer une contribution par une hausse objectif est d'asseoir le financement du fonds de lutte contre les addictions, qui est indispensable, sur les fabricants de tabac et d'éviter les contentieux liés aux difficultés de répercussion de la contribution. Ce nouvel équilibre

de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux départements par la loi de finances initiale pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l'État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ; l'alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO. Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l'APA (allocation personnalisée fait semblant de considérer que l'intention initiale du législateur était de ne vouloir compenser par ces mesures que les revalorisations exceptionnelles du RSA. Il n'en est rien

Au final, l'article 64 n'a pour seule finalité que de lier les trois recettes mentionnées au RSA, dans l'intention évidente de récupérer lesdits financements dans l'hypothèse d'une recentralisation du RSA.

compensation péréquée (DCP), la hausse du taux plafond des droits de mutation à titre onéreux et le fonds de solidarité en faveur des départements. Ces revalorisations exceptionnelles sont intervenues entre 2013 et 2018,

et des employeurs à la modulation au titre d'autres critères, y compris la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH). Le même critère a été retenu pour la modulation de la contribution due par les employeurs publics au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Les minima sociaux sont indexés sur l'inflation. Les retraites en deçà de 2 000 euros ne seront pas concernées par cette mesure de revalorisation maîtrisée, dont vous avez

par les économistes ou par les organisations syndicales. Au total, le montant moyen de la prime d'activité est passé de 159 euros en 2017 à 190 euros en 2020.

de l'article L. 432-1 du code des assurances, « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France

vote. Monsieur le rapporteur général,

Cet article pose un nouveau jalon pour davantage d'ambition et de cohérence avec l'accord de Paris sur le climat et l'engagement de l'Union européenne de supprimer les subventions aux énergies fossiles d'ici à 2020.

dans le code des assurances par l'article 68 : il faut s'assurer qu'aucun projet permettant d'augmenter la durée de vie ou la capacité de production d'installations existantes, au nom de la « réduction de l'impact environnemental » d'une centrale à charbon, ne puisse être soutenu par la puissance publique des garanties à l'exportation.

Or de nombreux industriels du secteur du charbon se cachent derrière cet argument de réduction de l'impact environnemental de centrales à charbon pour entreprendre des travaux permettant, en fait, de prolonger la durée de vie de celles-ci ou d'augmenter leur capacité de production. En adoptant cet amendement, nous pourrons y remédier.

pour s'assurer qu'aucun projet permettant d'augmenter la durée de vie ou la capacité de production d'installations existantes au nom de la « réduction de l'impact environnemental » d'une centrale à charbon ne peut être soutenu par la puissance publique à travers des garanties à l'exportation.

Nous proposons d'élargir les exclusions des soutiens au secteur du pétrole et du gaz à travers les garanties publiques au commerce extérieur. Il s'agit d'exclure tout soutien à la recherche, à l'exploitation ou à la production de nouveaux gisements d'hydrocarbures, ainsi qu'à toutes les infrastructures directement liées, notamment les infrastructures de transport. Dès lors, tout soutien aux projets liés au torchage de routine ou aux hydrocarbures non conventionnels serait exclu de fait.

ce sujet à bras-le-corps. En attendant, nous devons lui expliquer un certain nombre de choses. Après avoir été le premier pays à interdire, progressivement, l'exploitation des hydrocarbures sur son propre territoire, par la loi du 30 décembre 2017 dite loi Hulot, la France ne peut plus continuer à utiliser l'argent du contribuable pour

à exclure le soutien aux projets liés à l'exploitation de sables bitumineux, c'est-à-dire de sables imprégnés de bitume, exploitation qui génère en moyenne de trois à cinq fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que celle du pétrole classique et a des impacts environnementaux désastreux.

c'est-à-dire en amont de l'octroi des garanties, quand elles sont en cours d'instruction. En effet, pour faire remonter des informations sur les impacts environnementaux et sociaux depuis les communautés directement concernées, il est nécessaire de connaître les projets en cours d'instruction avant qu'une décision soit prise par la commission des garanties.

-sont vitales pour la viabilité économique de certains projets de recherche, d'exploitation et de production. Entraver leur financement risque donc de bloquer ce secteur, qui est absolument indispensable pour atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique au-dessous de 1,5 degré d'ici à la fin du siècle.

rempli : soit une baisse significative de leurs ressources, soit une augmentation importante de leurs charges. Il s'agit non pas de modifier l'enveloppe, mais d'offrir de la souplesse dans son affectation.

opérationnalité effective dès le début de 2020, conformément aux conclusions de la conférence du logement en outre-mer. Nous proposons donc d'insérer le texte rédigé par le Gouvernement dans le code de la construction en complétant son article L. 861-6.

consiste à aligner intérêts économiques et avancées écologiques. Cela vaut notamment pour l'économie circulaire, au sein de laquelle les agents jouent un rôle clef au tout début de la chaîne du tri. Il s'agit donc de mieux récompenser les comportements vertueux pour la collectivité. Aujourd'hui, de nombreuses communes françaises réfléchissent à mettre en place une part incitative dans leur fiscalité relative Elles rencontrent cependant de nombreuses difficultés organisationnelles, qui diffèrent d'un territoire à l'autre. Il convient donc à l'autre. Il convient donc de faciliter la mise en place de la part incitative en permettant aux structures qui le souhaitent de ne développer cette part que sur certaines parties de leur territoire en se fondant sur des critères objectifs liés aux caractéristiques des zones. Il s'agit de laisser aux territoires plus de souplesse pour expérimenter et trouver la solution la plus adaptée à leur réalité. est l'objet de cet amendement dont l'adoption permettra aux collectivités d'instituer une tarification incitative, afin d'encourager les agents à mieux prendre en compte l'importance du geste de tri. Quel est l'avis de la commission ?

d'une tarification incitative en matière de déchets, avec l'objectif que 15 millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025. Force est de constater que l'objectif est aujourd'hui loin d'être atteint. Pourtant de nombreuses grandes agglomérations françaises réfléchissent à la mise en place d'une part incitative dans leur fiscalité déchets. Elles se heurtent néanmoins à de nombreuses difficultés liées aux caractéristiques de leur territoire : formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, centre urbain extrêmement dense,

au regard de la récente décision de justice d'un tribunal administratif. C'est pourquoi cet amendement vise à sécuriser les redevances, notamment les redevances incitatives, en retenant l'analyse de la Cour de cassation.

Un régime dérogatoire permet aux intercommunalités qui ont transféré ces compétences à un syndicat de prélever elles-mêmes la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour le compte du syndicat. Ces dernières ont même une incitation à le faire, car elles peuvent alors intégrer ces recettes dans le calcul de leur coefficient d'intégration fiscale (CIF), donc bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement majorée. Or cette situation est source de confusions sur le terrain et crée un manque de visibilité globale pour les syndicats et les collectivités. Ainsi, une communauté de communes peut être amenée à défendre une redevance attaquée en justice, alors que celle-ci a été calculée par le syndicat. Faire face à ces complications implique un dialogue permanent entre le syndicat qui assure la collecte et la trésorerie des collectivités qui prélèvent la redevance. Or force est de constater que ceux-ci ne disposent pas nécessairement des moyens humains nécessaires. Cette lourdeur administrative est amplifiée, lorsque les collectivités concernées mettent en place la tarification incitative en vue de réduire les déchets sur leur territoire. En effet, cela complexifie encore le calcul de la redevance et les relations avec les habitants. Cette situation nuit au développement de la tarification incitative, qui est pourtant un outil essentiel pour réduire les déchets résiduels. Pour simplifier la mise en place Pour simplifier la mise en place de la redevance et favoriser la tarification incitative, sans pénaliser les collectivités qui bénéficient d'une dotation majorée en intégrant la fiscalité relative aux déchets dans leur coefficient d'intégration fiscale, il convient d'autoriser ces collectivités à intégrer ces recettes

théoriquement, il ne fait que substituer une ressource à une autre, c'est-à-dire attribuer aux communes de la taxe foncière à la place de la taxe d'habitation ; or, lorsque l'on en mesure les conséquences

Il aurait ainsi des effets paradoxaux. Ainsi, un EPCI qui se serait dessaisi de la gestion des déchets auprès d'un syndicat en lui confiant la perception des recettes associées serait considéré comme mieux intégré qu'un EPCI qui aurait laissé la compétence de gestion des déchets et les recettes associées aux communes. À notre sens, cela peut introduire une rupture d'égalité.

pour faire avancer la réflexion et apporter une réponse, car cette situation pose de véritables problèmes, notamment dans les intercommunalités qui confient à d'autres le soin de ramasser les déchets.

La Guyane est en effet le seul département où le permis de chasser n'est pas instauré. La mise en place de ce dernier, prévue par la loi relative à l'égalité réelle outre-mer, permet d'assurer une formation des chasseurs et d'améliorer le contrôle de la circulation des armes à feu. feu. Pour la Guyane, c'est un enjeu. Néanmoins, les coûts induits par les prestations liées au permis de chasser- droits de formation initiale, d'examen, de délivrance initiale, de renouvellement -risquent de constituer un facteur limitant, en particulier pour les populations autochtones, qui tirent traditionnellement leur subsistance de la chasse.

M. Maurice Antiste. Cet amendement a pour objet de maintenir en 2021 la contribution à l'audiovisuel public à son niveau de 2019, soit 139 euros et et 89 euros outre-mer, en augmentant son tarif de un euro en 2021 par rapport à celui de 2020 et en maintenant son indexation sur l'indice des prix à la consommation.

article. Les règles européennes plafonnent à 7 % la proportion de biocarburants de première génération pouvant être incorporés dans les carburants. L'objet de ce plafond est d'éviter les conflits d'usage entre l'alimentaire et le non-alimentaire. les biocarburants dits de seconde génération font l'objet d'une obligation d'incorporation fixée dans le code des douanes et d'une incitation fiscale. Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'augmenter en 2021 les objectifs d'incorporation d'énergies renouvelables dans la filière essence. il encourage en particulier l'incorporation, au-delà de 7 %, de composés dits « égouts pauvres », qui sont des résidus issus de la production de plantes sucrières. Or, contrairement à l'objectif fixé, cette disposition risque d'entraîner un conflit d'usage avec le secteur agroalimentaire, en particulier avec les producteurs de levure, qui dépendent en grande partie des approvisionnements en coproduits sucriers. Nul besoin d'expliquer les utilisations traditionnelles pour la fabrication de produits emblématiques de notre gastronomie, comme le pain, le vin, ou encore la bière. De nouveau, le développement des carburants dits alternatifs ne va sans poser de nombreuses questions. À l'heure où l'artificialisation des sols gagne chaque jour du terrain

sur lequel la vérité commande de dire que je manque d'éléments de réponse, mais il me semble que ce point avait également été pris en compte par le ministère technique. La parole est à M. René-Paul

faite. Lorsque l'on transforme la plante en entier, on arrive à la fois à nourrir les hommes et à trouver des produits biosourcés qui permettent de pratiquer la biochimie à la place de la pétrochimie.

accordé aux coproduits sucriers, c'est-à-dire à 0,5 % de l'énergie contenue dans les essences à partir de 2021. La production de bioéthanol étant déjà très dépendante de l'importation de coproduits sucriers, il n'est pas souhaitable d'augmenter cette dépendance démesurément. De leur côté, les producteurs de produits alimentaires, tels que la levure, ont besoin de ces coproduits sucriers. Une trop forte exonération sur ces produits entraînerait leur détournement vers la filière du bioéthanol, au détriment de la filière alimentaire.

à 0,4 % de l'énergie contenue dans les essences à partir de 2021. Quel

Le tallol est un coproduit de la pâte à papier, disponible en quantité limitée, valorisé depuis plus de 90 ans en substance chimique d'origine végétale et renouvelable dans des produits de la vie courante : pneus, adhésifs ou autres.

vise à abaisser le seuil maximal de contribution du tallol de 0,6 % à 0,1 % pour atteindre les objectifs d'incorporation des biocarburants dans la incitative relative à l'incorporation de biocarburants (Tirib). Le seuil de 0,6 % représente un volume d'environ 250 000 tonnes de tallol par an, soit plus du tiers de la ressource européenne, évaluée à environ 650 000 tonnes. L'industrie française de la chimie biosourcée utilise plus de 100 000 tonnes de tallol chaque année. Abaisser le taux maximal d'incorporation à 0,1 % permettrait d'assurer le maintien des activités de cette filière. Par ailleurs, il me semble plus judicieux de favoriser la valorisation matière des résidus et des coproduits plutôt que leur valorisation énergétique. Cet amendement est à visée préventive. À ce préventive. À ce jour, le tallol n'est pas utilisé dans la production de biodiesels en France, mais il est la seule matière première d'origine renouvelable

Cet amendement tend également au retrait du seuil maximal de contribution du brai de tallol, afin de rationaliser son traitement fiscal, cette matière première n'ayant pas d'utilisation concurrente à la valorisation énergétique.

pour la croissance verte, l'article L. 100-4 du code de l'énergie prévoit une multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable livrée par les réseaux de chaleur à l'horizon 2020. Or on dénombrait 13 370 kilotonnes équivalent pétrole de chaleur en 2017, alors que l'objectif est de 19 732 en 2020, selon le ministère de la transition écologique et solidaire. Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la biomasse, au moyen de l'exonération facultative de TFPB et de CFE qui est

1451 et suivants du code général des impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse. En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l'article 1382 et à l'article 1451 ne s'appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale mise en oeuvre par l'administration centrale a d'ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s'exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s'agit d'une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants. Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics. Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l'énergie elle-même.

Exonérer les installations de méthanisation non agricoles va très au-delà de l'objectif du dispositif en vigueur, qui est de soutenir la méthanisation agricole. Cette évolution conduirait à accorder une subvention injustifiée à des installations industrielles et à certains géants du secteur. L'efficacité de cette mesure, qui n'est ni chiffrée ni documentée, nous semble

une fiscalité incitative en direction des méthaniseurs non agricoles, qui sont utiles pour valoriser à des fins de production d'énergie les biodéchets des ménages et des professionnels.

dans beaucoup de secteurs. Le lait est un sous-produit de la méthanisation. Pour ma part, je préfère que l'on permette aux agriculteurs français de continuer à trouver un revenu complémentaire

Au lieu de compter sur la PAC, ils ont financé une partie de leur agriculture avec des subventions environnementales pour le solaire et la méthanisation.

en créant un signal-prix sur l'amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s'agit donc de placer le signal-prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l'objectif de division par deux du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement.

qui a été présenté précédemment. Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe- les assujettis resteraient les exploitants -, une telle mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal-prix voulu par le Gouvernement sur l'élimination des déchets, qui justifie l'augmentation de la TGAP en discussion dans le présent projet de loi de finances. En effet, avec une telle disposition, l'élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manoeuvre. Cela permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l'élimination des déchets sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.

Mme Viviane Malet. Les installations de stockage souhaitant bénéficier du taux réduit de TGAP stockage pour la valorisation à 75 % du biogaz capté vont devoir effectuer un mesurage direct des volumes de biogaz captés Or cette prescription est impossible à mettre en oeuvre dans les délais prévus par la loi. En effet, la plupart des instruments qui sont actuellement homologués sur le marché européen ne sont pas adaptés au mesurage du biogaz des installations de stockage, en raison de la composition hétérogène et du caractère corrosif

Toutefois, le dispositif du chèque eau calqué sur celui du chèque énergie n'est pas prévu. Cet amendement vise donc à intégrer les dépenses d'eau potable aux dépenses prises en charge par le chèque énergie.

Il s'agit de taxer les plastiques qui ne sont pas recyclés du fait de l'absence d'une filière. Le montant de cette taxe serait défini par un décret précisant aussi les dérogations sanitaires, médicales, alimentaires, et liées à l'isolation thermique ou électrique. Quel est l'avis de la commission ?

la croissance verte a fixé des objectifs précis et ambitieux. Je pense à la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de 50 % de la consommation d'énergie finale, à l'augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie ou à la rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017. Cela fait beaucoup. Cependant, force est de le constater, le risque que ces objectifs nationaux ambitieux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, en raison à la fois des prix bas de l'énergie et du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique. Cet amendement vise donc à faire des contrats de transition écologique un véritable dispositif ambitieux de début de déploiement de stratégies de transition écologique dans l'ensemble des territoires.

et d'édition de ces tarifs par le ministre chargé du budget, dans un objectif de fiabilisation des données nécessaires aux redevables pour l'établissement de leurs factures. Il vise, en avançant la date des opérations, à permettre une vérification du montant des tarifs avant leur entrée en vigueur pour éviter aux opérateurs l'envoi de factures rectificatives, au détriment des redevables réels de ces taxes. Cet amendement tend à modifier également les dispositions relatives à la substitution d'un syndicat aux communes dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants pour la perception de la taxe sur la consommation finale d'électricité. Il prévoit que la détermination du nombre d'habitants de la commune se fasse au 1 janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est perçue. La parole

Madame la secrétaire d'État, nos départements assument des compétences sociales représentant entre 50 et 60 % de leur budget de fonctionnement.

Malgré cela, ils ont dernièrement décidé, sans intervention du législateur et de l'État, de créer un fonds de solidarité et d'investissement interdépartemental, dans l'objectif de pratiquer une politique d'investissement permettant de renforcer la solidarité entre les territoires. Souvenez-vous également que nos départements doivent prendre en charge les dépenses extraordinairement lourdes pour accueillir les jeunes migrants, alors que la politique migratoire relève de l'État. Aussi, quand le Gouvernement dépose subrepticement à l'Assemblée nationale un amendement sur le projet de loi de finances pour 2020 visant à ponctionner les ressources des départements franciliens au profit de la Société du Grand Paris (SGP), permettez-nous d'être surpris, voire furieux Ce seront en fait 75 millions d'euros en 2020, puis 60 millions d'euros les années suivantes qui serviront à financer les engagements de l'État dans le domaine des transports inscrits dans le contrat de plan État-région 2020-2022. Je soutiendrai donc sans réserve les amendements tendant à supprimer l'article 72 . Mais permettez-moi cependant d'émettre un regret, celui que la commission des finances du Sénat ait jugé irrecevable mon amendement relatif aux ressources de la SGP. Je n'ignore pas Je n'ignore pas que le Grand Paris Express est un projet structurant, par conséquent coûteux, financé par l'emprunt. C'est pourquoi je proposais de porter de 15 % à 30 % le taux de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, créée l'an dernier sur l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale, Joël Giraud, et du député Gilles Carrez. constituait une alternative au prélèvement sur ressources des départements que vous nous imposez et aurait permis de faire supporter une charge relativement modeste aux touristes, qui bénéficient indiscutablement des infrastructures des transports franciliens.

Gouvernement, départements d'Île-de-France et région -sur un projet avec un réseau et des gares, qui ne satisfaisait pas tout le monde, mais qui était un compromis, ainsi que sur son financement. Le financement est assuré par les contribuables des huit départements

que l'on puisse prendre le temps de réactualiser le chiffrage et de voir ce dont on a besoin pour l'avenir. Je ne peux pas croire qu'il soit tellement urgent de décider quelque chose qu'il faille en passer par un moyen comme celui-là.

L'an dernier, ici même, la majorité sénatoriale a refusé un amendement visant à entériner la péréquation interdépartementale en Île-de-France à l'exception de Paris, alors même que tous les présidents

deux ou trois arguments. M. Léonhardt se demande comment justifier la contribution de l'ensemble des départements franciliens, alors même que le Grand Paris Express concerne quasi exclusivement les territoires de petite couronne et que ces investissements pharaoniques, évalués selon lui à 42 milliards d'euros, vont amputer durablement la modernisation du réseau existant. Pour que l'ensemble des Franciliens puissent bénéficier de cette nouvelle infrastructure, il sera indispensable que les usagers de la grande couronne puissent rejoindre ce nouveau réseau en RER dans des conditions normales, ce qui n'est absolument pas pris en compte actuellement. Le réseau RER, quand il de l'implosion, et les reports d'usagers de la route vers le RER qui découleront de la mise en place de la zone à faibles émissions d'ici à 2030 sont extrêmement préoccupants par la suite. Il convient donc,

Alors que le Gouvernement a lancé cette année une vaste réforme de la fiscalité locale qui affecte notamment les recettes des départements, il semble peu judicieux d'opérer un prélèvement additionnel sur les DMTO des départements franciliens. En outre, cela constituerait un précédent malvenu, alors que les départements ont besoin de temps pour s'adapter au nouveau schéma plus centralisé de leur financement.

il me semble que le Gouvernement témoigne d'un manque de respect envers le Parlement et les élus locaux en introduisant des mesures à la dernière minute relatives aux finances des collectivités, sans aucune concertation

Ces infrastructures vont faire évoluer la valeur des biens. Nous le savons tous, à partir du moment où l'on est à proximité d'une station de métro directement reliée au centre de Paris, on constate une appréciation

de récupérer cette survaleur liée au bénéfice de l'infrastructure et, ce faisant, vous désintéressez les départements du produit fiscal de leur propre dynamique urbaine.